Il est défendu.

Monsieur Laménie,

exceptionnelle, La loi du 16 mars 2015 a permis de faciliter la création de communes nouvelles en instaurant notamment un pacte financier garantissant pour les

je vous remercie